je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour vous présenter avec Olivier Dussopt les principales mesures de ce paquet pouvoir d'achat, qui comporte un projet de loi et un projet de loi de finances rectificative. Son objectif- je n'aurai de cesse de le rappeler au Sénat, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale -est de protéger nos compatriotes face à l'augmentation des prix sans équivalent depuis plusieurs années

et de l'électricité n'ont jamais été aussi élevés, il nous paraît essentiel, avec le Président de la République et la Première ministre, Élisabeth Borne, de maintenir le gel du prix du gaz

Nous avons par ailleurs trouvé un compromis à l'Assemblée nationale sur le fioul. Des députés d'autres groupes que le nôtre ont insisté sur la nécessité de mieux prendre en compte le coût supporté

pour tous nos compatriotes qui utilisent ce combustible pour se chauffer, tout en prenant aussi des mesures pour accélérer la transition et permettre à chacun de changer sa chaudière. Mais, comme un appareil ne peut pas se changer en deux semaines, nous avons accepté cette

Je veux redire mon opposition à toute nouvelle taxe dans notre pays, pour des raisons très profondes. En France, dès qu'une

Une taxe n'est pas une réponse à la situation économique de notre pays. Par ailleurs, taxer les entreprises nationales n'est pas la meilleure manière de renforcer notre économie, notre capacité à créer de la richesse et des emplois.

J'estime donc que nous devons tenir notre ligne, qui est aussi l'une des lignes directrices de la majorité : baisser les impôts, et ne pas considérer les taxes comme la solution aux difficultés des Français. aux difficultés des Français. Vous pouvez vous faire plaisir en réclamant des taxes, mesdames, messieurs les sénateurs. Je préfère faire plaisir à nos compatriotes en obtenant des remises qui vont directement dans leurs poches, plutôt que dans celles du Trésor public ! Cela restera ma philosophie et ma ligne de conduite.

Les textes que nous vous présentons proposent également des crédits pour reprendre à 100 % le contrôle de notre service public de l'énergie. EDF est un outil industriel fondamental pour l'approvisionnement énergétique et la souveraineté de notre pays. Mais l'entreprise fait face à des défis de modernisation importants : augmentation de la demande d'électricité, impératif de produire une énergie décarbonée, nécessité absolue de relancer le programme nucléaire ; le Président de la République a proposé à Belfort la construction de six nouveaux réacteurs EPR. Pour cela, nous avons besoin d'une unité de commandement totale sur EDF. Tel est l'objectif

pour les députés de la majorité, pour ceux qui refusaient la dérive de nos comptes publics et pour les ministres au banc du Gouvernement. Nous avons réussi à maintenir le cap. Nous sommes entrés avec 20 milliards d'euros de propositions d'aides pour nos compatriotes.

Le texte issu de l'Assemblée nationale a été enrichi durant son examen en commission. Je tiens avant tout à saluer la qualité de ces travaux, en précisant d'emblée que nous ne proposerons pas de revenir sur la plupart des modifications apportées en commission ; celles-ci améliorent très nettement le texte qui vous a été transmis.

Cette mesure exceptionnelle de pouvoir d'achat, que nous reconduisons pour la troisième année consécutive, concerne les salariés percevant moins de trois fois le SMIC, et ce jusqu'à la fin de l'année 2023. Nous avons aussi souhaité, en particulier après l'avis du Conseil d'État, créer un nouveau dispositif, pérenne celui-là, de partage de la valeur pour toutes les entreprises et tous les salariés, sans plafond de rémunération, assujetti au régime fiscal et social de l'intéressement. La commission des affaires sociales a fait le choix de le maintenir jusqu'au 31 décembre 2023 et d'en réserver ensuite le bénéfice aux seules entreprises de moins de cinquante salariés.

que cette exonération de cotisations sera intégralement compensée à la sécurité sociale par l'État, comme j'ai eu l'occasion de le dire devant l'Assemblée nationale. L'article 3 du projet de loi loi vise à faciliter le recours à l'intéressement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Notre objectif est de lever un maximum de blocages identifiés comme étant des freins au développement et au déploiement des accords d'intéressement. Nous accueillons très favorablement l'ajout de la commission, qui prévoit de réduire à quatre mois la durée maximale de la procédure d'agrément des accords de branches relatifs au dispositif de partage de la valeur. J'aurai toutefois l'occasion de vous proposer un amendement visant non pas à modifier l'économie générale du texte adopté par la commission, mais à préserver les seuls délais d'opposition

Je proposerai de le réintégrer. Il concerne la restructuration des branches professionnelles disposant de minima conventionnels durablement inférieurs au niveau du SMIC.

Je ne reviens pas sur l'article 15, qui prévoit les modalités de réembauche de salariés dans le cadre de la réouverture provisoire de la centrale à charbon de Saint-Avold. Je précise néanmoins

nous avons une troisième divergence, sur laquelle le Sénat, le Gouvernement et l'Assemblée nationale peuvent, me semble-t-il, travailler. La commission des affaires sociales a adopté un dispositif d'exonération forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires, dont le coût, pour une déduction forfaitaire de 50 centimes par heure supplémentaire,

le taux d'inflation devrait atteindre au moins 5,5 %, un niveau que la France n'avait pas enregistré depuis 1985. Nous avions collectivement fini par oublier les conséquences d'une forte inflation. Mais elles se rappellent brutalement aux Français, qui voient grimper en flèche le coût de la vie dans tous les territoires.

Or, loin d'y répondre, nombre d'articles du projet de loi transmis au Sénat la semaine dernière formaient un ensemble hétéroclite, ne présentant qu'un lien ténu avec l'enjeu de préservation du pouvoir d'achat des ménages. Notre commission a souhaité modifier le texte en partant d'un principe simple : apporter une réponse immédiate et concrète aux difficultés de nos concitoyens face à l'inflation, tout en privilégiant à cette fin la valorisation du travail.

Cette même approche nous a conduits à introduire un article 1, qui prévoit une réduction de cotisations sociales patronales sur la majoration de salaire au titre des heures supplémentaires. Car, pour que les salariés qui le souhaitent puissent récolter les fruits de leur travail, il faut que leur employeur soit en mesure de les payer. Dans un esprit de responsabilité pour nos finances publiques, l'article laisse au Gouvernement le soin de fixer par décret le montant de la réduction. L'allégement des cotisations sociales des indépendants, prévu à l'article 2, s'inscrit lui aussi dans une logique de soutien au pouvoir d'achat des travailleurs, pour un gain de l'ordre de 550 euros par an au niveau du SMIC. La commission a tenu à mieux encadrer le dispositif, à en corriger les imperfections et à en garantir la pérennité, sans oublier le cas spécifique des micro-entrepreneurs, qu'a abordé M. le ministre. Je regrette toutefois l'effet Je regrette toutefois l'effet de seuil lié à la forte augmentation du taux de cotisation prévu par le Gouvernement, entre 17 000 euros et 25 000 euros de revenus. Ce n'est pas de nature à inciter au travail. Du reste, les travailleurs indépendants ne percevront les frais d'une telle mesure qu'à compter du début de l'année 2023. Cette échéance est bien lointaine au regard de l'urgence de la situation. situation. L'article 5 prévoit une revalorisation de 4 % des prestations sociales au 1 juillet. Je le rappelle, il ne s'agit que d'une avance sur la revalorisation prévue par la loi au 1 janvier ou au 1 avril 2023. un soutien non négligeable sera apporté notamment à nos aînés, dont le pouvoir d'achat s'est particulièrement érodé au cours des dernières années, du fait des différentes mesures de sous-indexation des pensions mises en oeuvre par le Gouvernement.

évoquer les autres prestations concernées. Il est permis de s'interroger- je pense que nous aurons l'occasion de le faire -sur l'uniformité de la revalorisation proposée, compte tenu de l'objectif de valorisation du travail affiché par le texte.

Dans le prolongement des mesures de simplification proposées, nous avons prévu également de raccourcir les délais d'agrément des accords de branche sur l'intéressement et la participation. Ceux-ci doivent être rapidement applicables, afin que les petites entreprises les utilisent pour développer l'intéressement. Nous avons introduit dans le texte une mesure de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, qui apportera un soutien immédiat aux salariés dont les revenus sont insuffisants face à la hausse des prix.

Dans ce contexte- j'insiste sur ce terme -, de nombreuses branches professionnelles présentent des grilles de minima salariaux dont les plus bas échelons sont dépassés par le SMIC. Afin d'éviter un tassement des rémunérations au niveau du SMIC, l'article 4 entend inciter les partenaires sociaux à se saisir de la question par le biais du processus de restructuration des branches professionnelles. Il introduit une confusion entre un chantier structurel, qui doit engager toutes les parties prenantes, et les réponses conjoncturelles qu'appelle la protection du pouvoir d'achat des Français. La commission a considéré que les partenaires sociaux d'une branche éprouvant des difficultés structurelles à négocier sur les salaires ne seront probablement pas sensibles à la menace d'une hypothétique fusion.

La commission a donc supprimé cet article. Elle a en revanche proposé, dans un nouvel article 4 , une accélération des délais pour l'entrée en vigueur et l'extension des accords portant exclusivement sur les salaires lorsque plusieurs revalorisations du SMIC interviennent dans l'année. Ce projet de loi sert par ailleurs de véhicule à plusieurs dispositions visant à remédier à certaines situations inéquitables. L'article 5 , inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, vient clore le long débat sur la déconjugalisation de dans lequel le Sénat a été précurseur, en particulier grâce à l'action de notre collègue Philippe Mouiller et à celle d'autres sénateurs. Le revirement du Gouvernement, dont nous nous félicitons, rend possible la mise en oeuvre de cette réforme au plus tard le 1 octobre 2023. Cette date semble un peu lointaine, mais elle peut se justifier par la complexité technique de l'opération ; nous aurons l'occasion d'y revenir. Un mécanisme transitoire protège les perdants de la réforme, en leur permettant de bénéficier de l'AAH sous sa forme actuelle, jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'allocation si cette modalité leur est plus favorable. Nous attendons encore des garanties du Gouvernement. Nous proposerons un certain nombre d'amendements sur les modalités d'application du mécanisme. En outre, nous avons souhaité donner une base légale à l'instruction ministérielle permettant aux retraités exerçant un mandat électoral local de constituer des droits à pension de retraite en contrepartie des cotisations qu'ils versent. Les élus concernés pourront ainsi bénéficier en toute légalité des prestations sans devoir liquider leurs droits auprès de l'institution Enfin, la commission a approuvé l'article 15, qui permet l'embauche de salariés pour la réouverture temporaire de centrales à charbon. Le cadre dérogatoire au droit du travail ainsi prévu permet de répondre à une situation inédite pour notre souveraineté énergétique tout en assurant une protection satisfaisante des salariés et de l'employeur concernés.

Messieurs les ministres, vous l'aurez compris, notre commission s'est saisie de ce texte de manière à la fois critique et constructive. J'espère que nos débats permettront de l'enrichir et que la suite de la navette nous permettra surtout de nous montrer à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Très bien ! La parole est à M. le rapporteur

pouvoir d'achat ont été examinés par la commission des affaires économiques. Alors que nous traversons une crise inflationniste inédite, mais prévisible, notre commission regrette le manque d'anticipation, d'évaluation et d'ambition du texte. Nous déplorons aussi des conditions d'examen précipitées. Le Gouvernement indique vouloir bâtir une nouvelle relation avec le Parlement ; ce n'est pas gagné ! Et ce n'est pas admissible Sur le volet énergie, notre commission a recherché un équilibre entre, d'une part, la législation d'urgence et, d'autre part, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété. Nous avons

De plus, nous avons associé les collectivités à tous les dispositifs pertinents, dont l'interruptibilité du gaz. Enfin, nous avons circonscrit le champ des méthaniers flottants et complété leur programme d'investissement, gage de leur acceptation.

Tout en déplorant vivement la méthode, nous avons aussi adopté la validation d'un recours contre l'évolution de l'Arenh sur le plan des consultations, pour éviter toute hausse des prix. Souvenons-nous : le 4 avril dernier, ces prix avaient atteint 3 000 euros par mégawattheure : un record ! Ces mesures techniques et ponctuelles

Cela étant, notre commission a décidé d'apporter son soutien à ce volet, qui repose sur un compromis entre l'État, les locataires et les propriétaires visant à partager les effets de l'inflation sur les loyers et éviter une trop forte augmentation des charges des 7,4 millions de locataires.

il s'agit évidemment d'un maximum, qui n'a rien d'automatique. Il soutient en outre les ménages les plus modestes en augmentant dans la même proportion et par anticipation dès le 1 juillet deux paramètres de calcul des APL, tout en relevant par décret de 4

La faible ambition du texte trahit le fait que le Gouvernement envisage le sujet du pouvoir d'achat surtout et avant tout comme un sujet de revenus, et rarement comme un sujet de prix. Notre commission s'est donc attachée à rehausser l'ambition du texte et à s'assurer de son caractère opérationnel pour tous les acteurs. C'est pourquoi nous avons prévu que tous les contrats d'assurance conclus à distance ou par voie électronique devront désormais pouvoir être résiliés électroniquement. Compte tenu de la force de frappe des assureurs, il n'y a pas de raison de prévoir un dispositif trop restreint., afin de ne pas pénaliser les petites entreprises qui n'auraient pas les moyens informatiques de développer une résiliation en ligne,

Nous avons donc consacré le principe de la résiliation à tout moment, après la première reconduction, des contrats de services de télévision et de vidéo à la demande. jugé que les banques devaient être davantage sanctionnées lorsqu'elles tardent à rembourser leurs clients victimes de fraudes. Le schéma graduel que nous proposons permettra de les inciter à limiter leur retard.

Je pense que le Sénat mérite l'écoute complète du ministre.

pour les quatre articles relevant directement de ses compétences. Nous exprimons cette validation dans un esprit de responsabilité, mais sans enthousiasme particulier. particulier. Ce texte, dont le pouvoir d'achat des Français est loin d'être la seule finalité, nous inspire malheureusement plusieurs regrets sur le fond et la forme. D'abord, nous avons collectivement déploré les délais particulièrement contraints dans lesquels le Gouvernement nous demande de légiférer, qui ne sont pas indiqués pour travailler sereinement.

Bien entendu, nous ne nions pas l'urgence qui s'attache à traiter plusieurs sujets incontournables, afin de protéger le niveau de vie des Français face à l'inflation et sécuriser notre approvisionnement énergétique, en vue des hivers incertains qui s'annoncent dans un contexte géopolitique qui l'est tout autant. Il n'empêche : ce projet de loi aurait pu et dû être mieux préparé.

Si nous sommes aujourd'hui dans une telle situation, qui nous oblige à augmenter la production de la centrale de Cordemais, chère Laurence Garnier, à redémarrer la centrale de Saint-Avold, mais aussi à mettre en place un terminal méthanier flottant raccordé au réseau national de distribution du gaz naturel, c'est bien parce qu'il y a eu un manque de vision stratégique à long terme en matière d'indépendance énergétique. Nous avons bien compris que, sur ce sujet particulier, chaque jour compte. Nous veillerons, dans l'intelligence de nos débats, chère Agnès Canayer, à tenir le calendrier. Au rang Au rang des décisions inopportunes, je mentionnerai bien entendu la fermeture de la centrale de Fessenheim et le manque d'anticipation du vieillissement de nos centrales nucléaires.

S'ajoute à ces décisions notre retard sur le déploiement des énergies renouvelables, en particulier en matière d'éolien marin et de photovoltaïque. Enfin, le projet de loi comporte à mon sens un angle mort majeur

Du reste, les amendements adoptés par la commission ont permis, d'une part, d'apporter des garanties complémentaires pour l'information du public, l'environnement et la santé s'agissant du raccordement du terminal méthanier flottant au Havre et de mieux encadrer la compensation carbone des émissions des centrales à charbon, et, d'autre part, d'améliorer la

Désormais, l'indice des prix à la consommation est estimé à 5,6 % à la fin de l'année 2022. Il est très important d'avoir en tête que nous sommes face à un choc d'offre. Ce choc d'inflation, à l'origine très concentré sur l'énergie, puis sur l'alimentation, s'est désormais diffusé à l'ensemble du système des prix des produits manufacturés, mais aussi sur les services, avec un début d'accélération de l'ensemble du système de prix. D'ailleurs, selon les travaux de l'institut Rexecode, si les prix devaient se stabiliser à leur niveau du mois de juin, le choc d'inflation pour la seule année 2022 représenterait, toutes choses égales par ailleurs, une charge de 66 milliards d'euros 66 milliards d'euros par rapport à 2021 sur le revenu des ménages, soit environ 1 000 euros par habitant. Ce montant représente aussi 43 % de la surépargne des années 2020-2021, qui se trouve réintroduite dans le circuit pour maintenir le niveau de dépenses des ménages. La politique que le Gouvernement mène depuis la fin de l'année 2021, à l'origine pour répondre aux conséquences de la reprise de l'activité à la suite du confinement et de la crise sanitaire, a amorti le choc en France. Alors que la moyenne pour l'ensemble de la zone euro est de 1 288 euros par habitant

Or l'on constate aujourd'hui que les gains de productivité sont très en deçà de la progression du salaire réel. En 2009, lors de la crise financière, la productivité a baissé, mais les salaires ont continué de progresser, et l'écart a été rattrapé ensuite par la mise en place du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Est-ce encore possible aujourd'hui ? Non, car l'état de nos finances publiques ne permet pas de créer un nouveau CICE. Par ailleurs, la prime peut créer un effet d'aubaine pour les entreprises. Au premier trimestre de l'année 2019, l'Insee relevait que le salaire moyen par tête avait augmenté de 2,7 %, mais seulement de 1,3 % si on y retranchait l'effet de la PEPA, soit un niveau de croissance inférieur au trimestre antérieur et au trimestre suivant, où la hausse était plutôt de 1,5 %. Les entreprises ont-elles les moyens de participer ? Compte tenu de l'évolution de la structure des coûts des entreprises, le niveau de résultat d'exploitation rapporté à la valeur de leur production recule,

les 10 % des ménages les mieux lotis face à ce choc subissent une inflation de seulement 2,5 %, là où les 10 % des ménages les plus exposés subissent une inflation de 8,5 %. Cet écart se justifie moins par les revenus que par les lieux

L'inflation se nourrit également de l'afflux de liquidités. À cet égard, la généralisation et la pérennisation d'une prime centrée sur le pouvoir d'achat contribueraient à autoentretenir l'inflation. C'est la raison pour laquelle la commission des finances a décidé de recentrer le dispositif pour en faire un véritable dispositif de soutien au pouvoir d'achat des plus modestes.

de la commission. En application de l'article 44, alinéa 6, du règlement, la commission des affaires sociales demande la priorité d'examen et de vote sur l'article 15, immédiatement après l'article 5 . Je suis donc

règlement. Monsieur le président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 36 de notre règlement et porte sur l'organisation des débats. Visiblement, le changement de méthode tant vanté par le Gouvernement s'est évaporé avec la canicule de ces dernières semaines.

du texte. À l'évidence, ce périmètre est assez élastique, pour ne pas dire très subjectif d'un point de vue politique. Ainsi, le

pas dire de consensus politique et que l'on prône le changement de méthode, force est de constater que le temps d'aujourd'hui est pire que le temps d'hier et que les débats dans l'hémicycle au grand jour n'ont plus d'importance à vos yeux ! Vous y préférez bien évidemment l'obscurité des de régler vos affaires, entre Gouvernement et majorité sénatoriale

le Sénat se prononce sur un projet de loi de protection du pouvoir d'achat face à une situation d'inflation galopante, dont la cause principale, géopolitique, serait exceptionnelle, voire temporaire. Or si le choc est bien exogène, la gravité de ses répercussions, notamment pour nos approvisionnements en énergie, découle d'abord du retard pris dans la transition énergétique.

Que les choses soient claires : la remise en service d'une centrale à charbon ou la mise en place de terminaux méthaniers ne peuvent pas être des réponses durables quand l'urgence est de sortir des énergies fossiles ! Par le maintien de notre dépendance au gaz et au pétrole, nous payons le prix le prix fort de la plus grande illusion de notre temps, celle d'une énergie abondante, sans impact et bon marché. Aujourd'hui, c'est une économie au service de la construction de la sobriété qui doit se mettre en place. Il nous faut prendre la mesure de la raréfaction générale des ressources, qui, associée au dérèglement climatique, entraîne une inflation tendancielle et engager enfin des politiques d'adaptation. Car les dérèglements climatiques, comme la sécheresse, provoquent régulièrement une hausse des prix. Ainsi, en Italie, le manque d'eau a détruit au moins un tiers de la récolte saisonnière de riz, de maïs et d'alimentation animale ; en Inde, les plants de blé sont si dévastés que le pays interdit toute exportation.

pouvant atteindre 10 % à 20 % du PIB mondial à la fin du siècle ». De plus, ce modèle économique, Karl Marx, épuise deux choses : le travailleur et la nature. Je m'en explique : un autre facteur d'inflation provient de l'anticipation spéculative des grands groupes- entre autres, ceux de l'énergie et du transport -, qui profitent de la crise pour réaliser des surprofits, auxquels ni le Gouvernement ni la droite n'ont l'intention de s'opposer, enclenchant la boucle profits-prix.

en déconnectant les augmentations de salaire de la hausse des prix. C'est ce découplage, entamé depuis le tournant de la rigueur, qui a dégradé durablement le partage de la valeur ajoutée. Alors que, depuis 2017, les réformes antisociales et les baisses des contributions des entreprises continuent de déformer le partage du PIB au détriment du facteur travail, l'inflation actuelle nécessiterait, pour ne pas aggraver la crise sociale, des mesures ciblées et durables de soutien, notamment pour les catégories populaires, puisque l'inflation les frappe plus du fait de la structuration de leur consommation et de la part de leurs dépenses contraintes préengagées. Au lieu de quoi, nous avons des primes ponctuelles, désocialisées, défiscalisées, asséchant le salaire socialisé- or c'est le seul qui soit générateur de droits contributifs

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout ça pour ça ! Alors que nos compatriotes voient le coût de la vie flamber, tandis que les salaires n'augmentent pas, que les collectivités subissent de plein fouet l'augmentation du prix de l'énergie, comme celle des matériaux, vous nous présentez aujourd'hui un projet de loi prétendument de « pouvoir d'achat », qui n'en a que le nom Face à la montée des prix de l'essence, des denrées alimentaires, des loyers et des transports, le Gouvernement a décidé de répondre par des mesurettes qui ne remettent absolument pas en question ses choix de fond : les cadeaux aux plus grandes entreprises. Faut-il vous rappeler que la France est la championne des dividendes en Europe,

Certes, c'est déjà ça, pourrait-on dire ... Il y a quelques avancées pour les Français, comme la revalorisation de 4 % des minima sociaux, des prestations sociales et la revalorisation de 3,5 % du point d'indice des fonctionnaires, qui était gelé depuis des années.

Elles sont notoirement insuffisantes. Selon l'Insee, elles ne permettront d'améliorer le revenu disponible des ménages que d'un point. Vous parliez d'un bouquet de mesures s'apparentant au « bouquet de la mariée ». Finalement, ce sera un bouquet de chrysanthèmes Vous vous entêtez dans la logique libérale du laisser-faire au bénéfice des entreprises en facilitant le versement de primes défiscalisées et exonérées de cotisations sociales. Avec ce système, les patrons seront incités à accorder des primes plutôt qu'à augmenter les salaires. Autant de manque à gagner pour les comptes de la sécurité sociale ! Il n'y a aucun changement de braquet dans la répartition des richesses. Il s'agit juste d'un tour de passe-passe qui prend tout

tel affaiblissement programmé des comptes de la sécurité sociale justifiera d'ailleurs demain votre volonté de réformer notre système de retraite et de réduire les droits des salariés à travers une future réforme de l'indemnisation chômage. La droite sénatoriale partage cette vision, puisqu'elle a introduit dans le texte un article 1 qui prévoit la défiscalisation et la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Même en cas de compensation des exonérations par l'État, vous privez en réalité les services publics de moyens. Pour ne donner qu'un exemple, alors que les hôpitaux sont contraints de fermer leurs services d'urgences faute de personnels, vous prévoyez d'amputer le budget de l'assurance maladie de 500 millions d'euros supplémentaires sur le dos des travailleurs indépendants. Ces mêmes hôpitaux devront également payer les 2 milliards d'euros de revalorisation du point d'indice des agents hospitaliers, quand les collectivités devront payer les 2,3 milliards d'euros de revalorisation du point des agents de la fonction publique territoriale.

! C'est vrai ! Cela ne vous fait pas plaisir, mais c'est la réalité ! Aujourd'hui, le sujet fait l'unanimité. Face à l'urgence sociale, les familles ne peuvent pas attendre le 31 octobre 2023. Il faut arrêter l'hémorragie à la Caisse

la sécurité d'approvisionnement en électricité ou le transport routier de marchandises semblent bien éloignées du pouvoir d'achat et ne vont pas réduire les factures des familles. Il nous faut des mesures structurelles fortes, comme l'augmentation des salaires et pensions, celle du SMIC à 1 500 euros, ou la revalorisation de 10 % du point d'indice des fonctionnaires. Nous avions de nombreuses propositions alternatives,

Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste refuse de soutenir des revalorisations inférieures à l'inflation financées exclusivement sur le dos de la sécurité sociale sans mise à contribution des entreprises et des revenus financiers.

protéger le pouvoir d'achat des Français. D'aucuns pourraient regretter qu'il ne l'améliore pas. Je regrette pour ma part que nous ne parlions pas plus volontiers de « pouvoir de vivre ». En cet instant,

Évidemment, les moyens dont dispose le Gouvernement ne sauraient contraindre les employeurs à une augmentation des salaires hors SMIC. Il s'agit là de les aider, en luttant contre l'inflation économique, mais également démagogique

nous pensons que l'intéressement comme la participation en entreprise doivent être encouragés, voire facilités. Si l'accord d'intéressement reste une condition pour accorder cette prime dans les entreprises de moins de 50 salariés, les contrôles allégés et la capacité de l'employeur à prendre un accord unilatéral sont bienvenus. Il serait préjudiciable de s'en passer. L'article 2 n'appelle pas d'observations particulières. Nous accueillons favorablement la baisse des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants. Sur l'article 3, qui tend à favoriser l'intéressement, notre commission a permis d'assimiler les périodes de congé paternité à une présence en entreprise pour son calcul. Elle a également limité à quatre mois la durée de la procédure d'agrément

L'article 5 prévoit la revalorisation par anticipation des retraites et des prestations sociales. Nous soutiendrons évidemment ces dispositions, mais je veux dire ici notre opposition à toute tentative d'une revalorisation au rabais, notamment pour le RSA. Précisons que le droit prévoyait ces revalorisations. Le Gouvernement permet de le faire par anticipation sans dépasser ce qui aurait été dû. C'est bien l'esprit du texte. Je termine par l'article 5 . Il s'agit là de mettre fin à une injustice sociale en déconjugalisant l'AAH.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, madame la présidente de la commission

C'est ce qui est proposé dans le paquet législatif « pouvoir d'achat et PLFR ». Les enjeux sont clairs : protéger le niveau de vie, soit le reste à vivre ; relancer la consommation ; faire face à une crise énergétique, également sans précédent, le tout dans un contexte géopolitique dramatique, avec la guerre en Ukraine. Mon groupe, le RDSE, souhaite d'abord souligner les points positifs du texte présenté par le Gouvernement, comme la revalorisation de 4 % des pensions de retraite et d'invalidité, des prestations familiales, des minima sociaux et des bourses étudiantes, ou encore la revalorisation du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % par décret. Tout cela constitue un coup de pouce notable et immédiat. Nous devons aussi souligner l'adoption de l'amendement au PLFR qui a permis de compenser la hausse du RSA par une dotation de 120 millions d'euros aux départements. un autre pour apporter de l'aide à certaines communes. Nous sommes plus réservés sur l'article 1. Une prime, c'est bien ; une augmentation de salaire, c'est mieux En effet, si 20 % des salariés en ont bénéficié, le versement moyen est de 546 euros, au lieu des 1 000 euros possibles jusqu'à maintenant. Alors, à quoi sert d'augmenter le seuil, sinon à se faire plaisir avec des effets d'annonce ? Sur le modèle de l'article 2, qui prévoit une exonération de charges pour les travailleurs indépendants, il aurait été préférable de pousser plus loin les exonérations de charges sociales ou de la contribution sociale

d'un côté, on accroît de 3,5 % les APL, et, de l'autre, on bloque à 3,5 % l'augmentation des loyers. Certes, on bloque, mais cela n'évite pas l'effet pervers mathématique Si le plus ancien groupe du Sénat ne peut pas se permettre d'emprunter l'expression « d'enfumage », chère à certains députés, il n'en pense pas moins ! Nous constatons que les 8 euros en moyenne gagnés grâce à la hausse des APL ne compenseront jamais l'augmentation des loyers. Par exemple, pour un loyer de 600 euros, pourra être de 21 euros. Je ne crois pas que l'effort profite à tous de la même façon. De plus, des locataires qui ne touchent pas d'APL et qui ne sont pas pour autant des nantis ?

les quatre centrales à charbon produisaient 1,3 % de l'électricité nationale et 30 % des gaz à effet de serre du secteur électrique ... Sans commentaire

Entre crise sanitaire, crise géopolitique, crise énergétique, les Français payent le prix fort. De nos débats et de nos votes dépend leur quotidien. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement, ayant confiné tout l'été, se trouva fort dépourvu quand l'inflation fut venue ! Pas un seul petit morceau de regain dans les hôpitaux. Il administre de la morphine au contribuable en famine. Ce projet de loi sur le pouvoir d'achat annonce un saupoudrage ponctuel et coûteux dans un contexte d'inflation historique et durable. Il ne réglera donc rien ! Vous nous demandez d'arroser d'une goutte d'eau la plante dont vous avez asséché le terreau en ayant voulu jouer au mariole avec votre politique du « quoi qu'il en coûte a laissé sous-entendre, à tort, une forme de générosité de l'État, alors que, Margaret l'a dit avant moi : « L'argent public n'existe pas ; il n'y a que l'argent des contribuables. » À l'épisode de l'argent magique succède désormais celui de l'appauvrissement tragique. Contrairement à ce que vous tentez de nous faire croire, la cause russo-ukrainienne est marginale dans l'explosion de l'inflation. Celle-ci a commencé début 2021, comme la conséquence directe des confinements, avec les dix-huit mois de restrictions et le recours massif à l'usage de la planche à billets par les banques centrales. Depuis, nous avons eu la hausse des prix de l'énergie, du prix à la pompe, des denrées alimentaires. Si vous ne voulez pas revoir les rues de France couvertes de « gilets jaunes » rouges de colère, il faut agir, et vite, monsieur le ministre Nous pourrions, par exemple, remplacer au moins 25 % du total de la prime de Noël et de l'allocation de rentrée scolaire par des bons d'achat fléchés exclusivement vers des produits fabriqués en France, soit 1,25 milliard d'euros pour l'emploi, sans aucune dépense publique supplémentaire. Le meilleur moyen de débloquer de l'argent pour nos compatriotes, c'est d'abord de ne pas leur prendre ce qu'ils ont gagné. Mettez un terme à votre racket fiscal envers ceux qui entreprennent, ceux qui travaillent et qui, donc, produisent de la richesse vous qui, par votre incurie énergétique, voulez rationner les Français en énergie, commencez par rationner l'État en impôts ! Sobriété bien ordonnée commence par soi-même, d'autant que l'année 2023 s'annonce. L'explosion de la dette va mécaniquement entraîner l'explosion des intérêts de la dette, qu'il nous faut payer chaque année. Ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros supplémentaires qu'il va vous falloir trouver. En augmentant les impôts ? Impossible, les Français ne le supporteraient pas ! En rognant sur les budgets des ministères ? À l'exception des budgets dédiés à l'immigration, ils sont à l'os ! De l'argent, il y en a, et beaucoup. Je vous propose de prendre d'urgence les mesures pour lutter contre l'assistanat, contre la fraude sociale, qui atteint 50 milliards d'euros, la fraude fiscale et ses 70 milliards d'euros, et, bien sûr, le gouffre de l'immigration, qui, sans parler du coût du sang, coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros aux contribuables français ! Avec 600 milliards d'euros de dette sous le premier quinquennat et 10 millions de Français qui survivent sous le seuil de pauvreté, réussir à s'en sortir, et seulement à s'en sortir,

Vous dépensiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, monsieur le ministre, renflouez maintenant

il faut une réponse systémique à la nécessité de rendre aux travailleurs et aux citoyens cette puissance d'agir que constitue la possibilité d'assurer sa subsistance, de consommer, de construire son quotidien, ainsi que sa place dans la société et sa protection sociale. Nous espérions donc dans ce projet de loi une valorisation du travail, une clarification de ce qu'est le travail et des droits qu'il apporte. Nous attendions des mesures permettant de consolider le salariat et notre système de protection sociale. Rien de tel dans ce texte, qui ignore la question salariale, pourtant au coeur de celle du pouvoir d'achat ! Je dirais même que la réponse systémique du Gouvernement vire au cynisme. Vous jouez de diversion au moyen de multiples mesures, dont certaines dépassent formellement le champ des affaires sociales, pour finalement aggraver la prédation à l'encontre de la sécurité sociale. Vous faites le choix délibéré d'un revenu désocialisé et défiscalisé. Et c'est sous la pression de la crise inflationniste que les travailleurs, pris à la gorge, se voient proposer la substitution de la prime au salaire, parallèlement à une modération du coût du travail, c'est-à-dire des salaires. Avec la prime de partage de la valeur, l'exceptionnel devient donc la règle. Cette prime pérennise en effet un dispositif facultatif, temporaire et discrétionnaire. Ainsi, le plafond de la « prime Macron » est augmenté pour atteindre 6 000 euros. Ce chiffre crée une diversion. Nous savons en effet que, malgré un plafond passé à 2 000 euros depuis sa mise en place en 2019, le montant moyen de cette prime n'a jamais dépassé 506 euros.

Monsieur le ministre, les Français ne demandent pas l'aumône. Ils demandent des salaires justes, une protection sociale de qualité et des conditions de travail dignes. Dans le même temps, et parce que cela va de pair, le Gouvernement continue à faire du dialogue social un simple décor en renvoyant les partenaires sociaux à un statut de figurants. En atteste son choix de faire mine d'inciter les branches à la négociation sur les salaires avec son article 4, qui ne constitue pas, à notre sens, un soutien suffisant aux revalorisations salariales. Si les travailleurs pauvres et les « premiers de corvée » sont ignorés ici, l'enjeu n'est pas seulement la modération salariale. Il s'agit aussi de programmer l'obsolescence du salariat et des protections qu'il apporte. L'intéressement croissant à l'épargne salariale voulue par le Gouvernement est de fait un dispositif d'évitement du salaire, ce qui participe de ce mouvement. Il donne le pouvoir à l'employeur de décider unilatéralement de mettre en place ce dispositif dans les entreprises de moins de 50 salariés, en cas d'échec des négociations ou en l'absence d'institutions représentatives du personnel. Le texte fragilise donc la sécurité sociale en la privant de ressources dans l'objectif, toujours, de relancer l'activité économique. Le patrimoine que constituent pour les Français les assurances sociales est en effet dilapidé par le Gouvernement depuis longtemps. Je pense au choix de faire porter sur la sécurité sociale la dette covid et au refus de compenser le trou creusé par les 2,8 milliards d'euros de mesures prises en réponse à la crise des gilets jaunes. La revalorisation exceptionnelle de 4 %, qui est une bonne chose, n'est par ailleurs pas suffisante pour améliorer le tableau de votre texte. Il faut la mettre à 10 % ... Elle ne fait qu'anticiper les revalorisations de droit commun prévues d'octobre 2022 à avril 2023, et elle ne suffira pas à compenser la forte augmentation de l'inflation, évaluée par l'Insee de 6 % à 7 % cette année. Au registre des déceptions, la majorité du Sénat emboîte d'ailleurs le pas à l'exécutif, puisque, peut-être inspirée par le choix de l'Assemblée nationale de mettre en place une monétisation des RTT menaçante pour les 35 heures, elle a décidé de baisser les cotisations patronales au titre des heures supplémentaires. Cette logique de fragilisation de la sécurité sociale est aussi à l'oeuvre avec la baisse pérenne des cotisations des indépendants. Pour un gain de 550 euros de revenus annuels, on sacrifie ainsi leur protection sociale. Cela confirme la marche vers l'ubérisation du travail, que nous dénonçons maintenant depuis plusieurs années. Vous refusez l'idée d'une grande conférence sur les salaires, qui aurait pour objectif d'amener les employeurs à augmenter les salaires. Et, dans le même temps, vous leur donnez les outils pour contourner le salariat., salariat., nous savons tous qui seront les perdants, et la grande idée de loi sur le pouvoir d'achat ne sera que le faux nez d'une stratégie de fragilisation du salariat. Cynisme toujours

Lemoyne. Monsieur le président, mesdames, messieurs les présidents de commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, mes chers collègues,

L'État a été là. Dès l'automne dernier, sans délai, le bouclier tarifaire était mis en place pour limiter la hausse des coûts de l'énergie pour les ménages, les petites entreprises et les petites communes.

ce projet de loi est à nos yeux trois fois nécessaire ; c'est pourquoi le groupe RDPI lui dira donc trois fois oui ! Oui, pour juguler l'inflation ! Je note à ce propos que les Français sont mieux protégés que les autres Européens. Oui, pour mieux protéger les consommateurs

que chacun puisse avoir un travail rémunérateur. La juste considération, c'est la juste rémunération, et non pas juste une rémunération. Alors, monsieur le ministre, nous serons à vos côtés pour défendre le pouvoir d'achat. Nous le serons aussi, tout au long des prochains mois, pour mener d'autres transformations, afin que chacun ait le droit de vivre dans la dignité ! La parole

La forte reprise économique au sortir des confinements a provoqué des tensions sur bon nombre de marchés, dont ceux des matières premières, des énergies, mais également des semi-conducteurs. Cette situation inflationniste a été encore aggravée par l'invasion russe de l'Ukraine. En entrant en confrontation avec l'Europe, la Russie bouleverse l'équilibre énergétique qui y prévalait. La France, qui compte pourtant parmi les pays les moins touchés par l'inflation, a vu le niveau général des prix augmenter de près de 6 % lors des douze derniers mois. Cette situation a de lourdes conséquences pour bon nombre de ménages, malgré les aides déjà accordées par l'État. Elle aura aussi, à n'en pas douter, de graves répercussions sur nos finances publiques, mais chaque chose en son temps. D'abord, l'urgence L'urgence, c'est de faire en sorte que le travail soit mieux revalorisé, en donnant pleine efficacité à la prime de pouvoir d'achat. J'estime cependant que celle-ci ne doit pas se substituer aux revenus et qu'un encadrement strict devra garantir que le recours à ce dispositif À ce titre, je défendrai plusieurs amendements tendant à simplifier cet outil mis à la disposition des entreprises pour le bénéfice des salariés, de manière à renforcer son efficacité. Le travail déjà effectué en faveur des professions libérales et des micro-entrepreneurs me paraît tout aussi essentiel. Notre pays a la chance de pouvoir compter sur des forces vives importantes et doit préserver son tissu d'entrepreneurs. La simplification du cadre juridique de l'intéressement est aussi à saluer. La souplesse jouera en faveur des salariés et des entreprises. Mais il est également très urgent, monsieur le ministre, de mener une réflexion avancée sur notre droit du travail. Celui-ci doit être simplifié et adapté aux enjeux du siècle. Il doit gagner en agilité et en flexibilité pour les évolutions futures. Nous serons au rendez-vous de ces discussions quand le temps sera venu. L'autre grand défi que la France et ses partenaires européens doivent relever est celui de la souveraineté énergétique. L'Europe est condamnée à la dépendance, dans la mesure où elle doit importer les matériaux nécessaires à la production de son énergie. Cette dépendance n'est pas incompatible avec sa souveraineté, à la condition que l'Europe parvienne à s'approvisionner auprès de sources diversifiées et sûres. Le gaz russe manquera cet hiver. Pour compenser, il convient notamment d'importer davantage de gaz naturel liquéfié. Ce dernier est cependant plus cher et la France devra se doter rapidement d'équipements nécessaires à son exploitation. Le parc nucléaire français ne suffira pas, en l'état, à subvenir à nos besoins. À ce titre, les évolutions concernant l'Arenh vont dans le bon sens. Le nucléaire est une chance pour notre pays ; il faut le préserver. Mais notre parc est vieillissant. Les investissements seront la clef de notre souveraineté énergétique. Le nucléaire, quelle que soit la forme qu'il prenne, (EPR) ou (SMR), restera un atout de transition, au même titre que les énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert, l'hydrogène vert, sous réserve que nous sécurisions notre approvisionnement en uranium. Certaines centrales à charbon devront malheureusement être réactivées. Cette situation ne saurait être pérenne. Nous devrons continuer de consolider notre souveraineté énergétique dans les années à venir, tout en respectant nos engagements dans la lutte contre le dérèglement climatique. La sobriété et l'efficience seront deux alliés majeurs grâce notamment à une plus forte décentralisation de la production et de la consommation des énergies renouvelables. Cela passera par l'innovation et la réindustrialisation,

Nous devons cependant garder à l'esprit que ces mesures, dans leur ensemble, auront de graves conséquences sur nos finances publiques. La France doit s'assurer de bâtir son avenir sur des bases solides. La parole

Il s'agit de réagir dans l'urgence à deux événements majeurs : la hausse brutale de l'inflation et les difficultés d'approvisionnement énergétique de la France. Mais, force est de le constater, le projet du Gouvernement repose essentiellement sur l'attribution ponctuelle de chèques, ce qui ne représente pas une politique en soi. Je m'attacherai à évoquer le volet social du projet de loi. Je note tout d'abord des mesures de pure communication, telles que le triplement de la prime dénommée « de partage de la valeur », mesure phare censée améliorer le niveau de vie des Français, son montant pouvant aller jusqu'à 6 000 euros dans certains cas. Toutefois, le montant moyen des sommes versées au titre de la prime Macron s'est situé autour de 500 euros, et cela n'a concerné que très peu de travailleurs : un actif sur cinq. même volonté d'affichage lorsque le Gouvernement appelle les branches professionnelles à négocier sur les salaires. L'article 4 n'était guère incitatif et était si peu approprié à la situation des très rares branches concernées que notre commission a décidé de le supprimer. Si nous ne pouvons qu'acquiescer aux aides ciblant certains publics- revalorisation anticipée des retraites, baisse de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants -, nous constatons également un saupoudrage de moyens, dont l'addition finit par grever de façon alarmante les finances de l'État.

Néanmoins, ils ont émis des propositions pour financer ces mesures, notamment par des économies importantes dans le fonctionnement bien trop lourd de nos administrations. Nous proposerons pour notre part, dans le projet de loi de finances rectificative, de lutter contre la fraude sociale par la mise en place d'une carte Vitale biométrique. Notre logique politique est claire : au lieu d'une politique de l'assistanat, nous souhaitons privilégier la solidarité et l'aide au travail. Nous pensons que le pouvoir d'achat doit garder son lien avec le travail et que celui-ci doit être privilégié par rapport à l'assistance.

notre rapporteur Frédérique Puissat, dont je salue la qualité du travail et l'investissement sur ce texte, a proposé d'alléger les cotisations sociales des entreprises d'au moins vingt salariés, renforçant ainsi l'attractivité du dispositif. par l'Assemblée nationale, nous avons obtenu du Gouvernement que des heures de RTT puissent être rachetées par les salariés souhaitant travailler plus pour améliorer leur pouvoir d'achat. Ces mesures devront être définitives, et non pas seulement provisoires, comme le souhaite le Gouvernement. Gouvernement. Notre commission a adopté un amendement permettant exceptionnellement le déblocage des sommes issues de la participation et de l'intéressement placées sur des plans d'épargne salariale. Cela permettra aux salariés de disposer d'un pouvoir d'achat immédiat, jusqu'à 10 000 euros, avant le 31 décembre prochain. De même, notre rapporteur a proposé d'assouplir les règles encadrant l'utilisation des titres-restaurant. Ceux-ci pourront être utilisés pour les achats alimentaires courants dans les commerces de détail et les supermarchés, ce qui répond à un vrai besoin. Ce sont autant de mesures qui auront un effet direct sur le pouvoir d'achat.

revalorisation ne soit pas supérieure à celle du point d'indice pour les fonctionnaires. En effet, nous ne pouvons pas adresser comme message aux Français que les revenus de l'assistance sont privilégiés par rapport aux revenus du travail.

et les associations : la déconjugalisation du mode de calcul de l'allocation aux adultes handicapés, à l'article 5 . Je me réjouis particulièrement de cette issue en tant que rapporteur de la proposition de loi que nous avions adoptée le 9 mars 2021, sur toutes les travées de notre Haute Assemblée,

À l'heure où le pouvoir d'achat des plus fragiles est particulièrement menacé, je pense que l'esprit de solidarité doit l'emporter sur les règles technocratiques. Je note d'ailleurs que nous sommes finalement parvenus à un accord sur ce dossier qui dure depuis des années et que l'édifice des minima sociaux ne s'est pas écroulé pour autant ! Encore reste-t-il à adapter le dispositif au cas par cas. Comme je l'avais souligné lors de l'examen de la proposition de loi, la déconjugalisation peut faire des perdants. Il s'agissait d'ailleurs de l'argument principal opposé à notre demande. Un mécanisme transitoire, permettant de conserver le bénéfice des règles de calcul actuelles dans les cas les plus favorables, a été trouvé. Je m'en réjouis. Toutefois, comme l'a indiqué notre rapporteur Frédérique Puissat, une précision est nécessaire pour les bénéficiaires de l'AAH qui se trouveront en situation de renouvellement de leurs droits. De plus, je regrette que cette déconjugalisation, pour des raisons techniques, ne puisse pas entrer en vigueur avant le 1 octobre 2023.

; je pense au grand sujet de l'évolution de la prestation de compensation du handicap (PCH). Ce n'est pas l'objet du présent texte, mais nous devrons engager des travaux dans les prochaines semaines sur ce sujet fondamental, pour une réforme globale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un contexte de forte inflation, d'explosion du prix de l'énergie et de hausse constante du coût de la vie, la préservation du pouvoir d'achat des Français est désormais plus qu'une boussole ; c'est un impératif ! Il faut entendre la détresse et, parfois, la colère de nos concitoyens. Difficulté à boucler les fins de mois, anxiété à l'idée de faire le plein de son véhicule, sacrifices au quotidien : nous ne pouvons pas rester sourds ni aphones face à ces situations compliquées. : le projet de loi pour la protection du pouvoir d'achat répond-il aux besoins des plus fragiles ? Va-t-il améliorer durablement les conditions de vie ou de survie des plus touchés par l'inflation ? La réponse est non ; durablement non ! Néanmoins, avec mes collègues de l'Union Centriste, nous sommes persuadés que les dispositions contenues dans ce projet de loi sont, quoi qu'il en soit, les bienvenues dans un contexte aussi difficile. Il ne s'agit pas de donner un blanc-seing au Gouvernement. Mais je crois que, dans cet hémicycle, nous devons faire primer le bon sens et l'intérêt général. À ce titre, nous saluons la revalorisation des minima sociaux, la résiliation facilitée des abonnements conclus par voie électronique, le plafonnement des loyers pour les ménages et, enfin, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés, qui reconnaît un statut pour l'adulte en situation de handicap. Mais qu'en est-il des aides ciblées, d'aider les Français en ayant le plus besoin ? On ne peut plus financer de manière aveugle des aides généralisées en continuant de creuser le déficit public, aides qui sont d'ailleurs souvent supportées par les collectivités. une question de justice sociale : les politiques publiques doivent cibler les plus fragiles pour les soutenir durablement. Je pense à nos aînés, à nos étudiants, aux familles monoparentales, aux classes moyennes, c'est-à-dire à ceux qui doivent payer toujours plus pour gagner de moins en moins. Ce texte est également l'occasion d'aborder l'enjeu de notre souveraineté énergétique. Une véritable course contre la montre s'engage pour éviter cet hiver des ruptures d'approvisionnement, en électricité notamment.

Saint-Avold ? Nous formulons deux voeux : une nouvelle méthode de travail et un cap stratégique qui redonnera confiance à nos concitoyens, à nos entreprises, à nos élus. Pour ce qui est de la méthode de travail, le quinquennat qui s'ouvre devait être celui de la coconstruction législative et d'un travail plus collaboratif avec le Parlement,

Qu'adviendra-t-il en janvier 2023 pour nos concitoyens, lorsque les remises sur le carburant ne seront plus appliquées ? Quelles garanties en matière d'approvisionnement en électricité pourrez-vous offrir aux entreprises qui envisageraient de s'installer en France ? Quelles réponses apporterez-vous aux collectivités qui s'interrogent sur la faisabilité de leurs projets d'investissement face à l'augmentation toujours croissante de leurs dépenses de fonctionnement et à la baisse de leurs recettes ? Ces questions concrètes appellent des réponses précises. La parole est à M.

M. Franck Montaugé. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en matière de logement et du point de vue des usagers les plus modestes, donc les plus touchés par l'inflation, les dispositions visant à contenir les hausses de loyers ne sont pas assez fortes. Nous proposerons un plafonnement à 1,5 % de l'IRL sur tout le territoire national. Pour mémoire, la diminution de l'APL vous a permis d'économiser 12 milliards d'euros lors du quinquennat précédent. Or les mesures que vous proposez dans ce texte représentent seulement 168 millions d'euros Disons-le sans ambages : les dispositions du titre II, relatives à la protection du consommateur, qu'elles portent sur la résiliation des contrats ou sur la lutte contre les pratiques commerciales illicites, bien qu'opportunes, sont de portée réduite. Nous vous proposerons par nos amendements de les améliorer. Les mesures du titre III, relatives à la souveraineté énergétique, pour autant qu'elles soient nécessaires, révèlent les faiblesses et les contradictions de la politique française La crise aura permis de mesurer l'attention qu'il faut en permanence porter à l'outil de stockage souterrain de gaz, outil stratégique s'il en est, dont la dimension de politique nationale a été oubliée ou mésestimée. En même temps qu'elle porte atteinte à la crédibilité de la parole publique, la nécessité de prévoir la réouverture de centrales à charbon pose pour nous la question des conditions sociales du réemploi et de la formation du personnel nécessaire. de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique confirment ce que nos rapports sénatoriaux récents ont mis en évidence : l'affaiblissement régulier d'EDF, jusqu'à sa mise en péril au regard des investissements considérables à financer dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie, que nous aurons à actualiser prochainement. En matière de climat, la France doit être au rendez-vous de ses engagements, après cinq années perdues et deux condamnations pour inaction climatique. Au-delà des évolutions nécessaires de l'Arenh qui figurent dans le texte et que nous soutiendrons, comme la limitation de volume à 100 térawattheures ou à 25 % de la production nucléaire annuelle, au prix actualisé de 49,50 euros nous demandons d'anticiper l'extinction et la suppression totale du mécanisme, tant l'Arenh s'est jusqu'ici révélé comme un instrument de pillage et d'affaiblissement d'EDF au profit de ses concurrents.

au Conseil supérieur de l'énergie (CSE) ni notifié formellement à la Commission européenne. Pourquoi, monsieur le ministre, avoir procédé de la sorte, en toute connaissance d'une aide d'État dont l'absence de notification fragilise aujourd'hui les fournisseurs alternatifs ? Il est urgent de reconsidérer,

nous demandons le vote d'une loi spécifique sur le projet industriel, social et environnemental d'EDF. En outre, le Gouvernement devra réussir le plus rapidement possible une réforme de structure des tarifs de l'électricité, qui doivent reposer sur les coûts complets de long terme de l'ensemble du parc de production. Au final, le présent texte sera insuffisant pour répondre aux besoins élémentaires de millions de Français. Le « pouvoir de vivre » de nos concitoyens sera au coeur de nos propositions dans les prochains projets de loi de finances. La parole

nous l'attendions, ce texte sur le pouvoir d'achat, promis depuis bien des semaines et enfin inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée, malgré des délais très courts pour son examen par le Sénat. Je voudrais rappeler que, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, 66 % des Français citaient la question du pouvoir d'achat comme l'enjeu principal de cette élection, selon le baromètre OpinionWay. Le Gouvernement nous présente donc, comme d'autres l'auraient fait d'ailleurs, un projet de loi censé atténuer les effets de l'inflation et de la crise énergétique tout en contenant les déficits publics.

Aussi, il faut pouvoir trouver la ligne de crête entre le soutien à ceux de nos concitoyens qui souffrent le plus de la situation actuelle et la nécessité de ne pas alourdir la dette publique pour préparer l'avenir et la nécessaire transition écologique, qui impose des investissements massifs. Alors, que nous propose le Gouvernement ? D'abord, un texte insuffisamment ambitieux, avec des mesures qui peuvent sembler anecdotiques au vu de la situation, comme la possibilité de résilier par voie électronique les contrats souscrits en ligne. Ensuite, un texte qui n'a rien de structurel : j'en prends pour preuve les mesures concernant le plafonnement de la hausse des loyers. C'est clairement ignorer les solutions de long terme qui favoriseraient la construction de nouveaux logements, alors que c'est bien le manque de logements qui explique aujourd'hui la tension sur les loyers. Enfin, un texte qui est en contradiction avec certaines de nos politiques publiques, particulièrement dans le domaine énergétique, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises. Nous légiférons aujourd'hui pour rouvrir les centrales à charbon après avoir décidé de les fermer et, surtout, après des années d'hésitations et de contradictions sur le développement du nucléaire ! Nous allons aussi importer des hydrocarbures après avoir abandonné la filière nationale et fragilisé les filières françaises décarbonées.

Restaurer la souveraineté énergétique de la France nécessitera d'être cohérent dans les choix effectués et, en l'espèce, nous pouvons regretter que cela n'ait pas été le cas ces dix dernières années.

Pourquoi pas ? Mais pour quoi faire ? Et pour changer quoi ? Cela ne répond pas aux difficultés du groupe, notamment au mur d'investissement auquel il doit faire face. Nous prônons depuis longtemps un énergétique décarboné autour du nucléaire, et ce dans un bouquet d'énergies. Le récent rapport d'information de nos collègues Gremillet, Moga et Michau a encore déploré l'affaiblissement de la filière, ainsi que ses perspectives très complexes. Il contient des propositions pour relancer l'énergie nucléaire et promouvoir l'hydrogène bas-carbone, dont le Gouvernement devrait s'inspirer. Nous prônons également le développement des énergies vertes : l'eau, le vent, le soleil, la biomasse, le biogaz. biogaz. Monsieur le ministre, mes chers collègues, rien ne doit être négligé pour atteindre la neutralité carbone. J'ai d'ailleurs présidé voilà peu la mission d'information sur la méthanisation. Nous avons, là aussi, des pistes utiles pour favoriser la transition et la souveraineté énergétiques si nous nous donnons les moyens de structurer la filière et de simplifier- je dis bien simplifier -l'ensemble des procédures. L'actualité nous l'impose plus que jamais. Au final, le texte que nous examinons aujourd'hui me paraît très décevant, même s'il comporte des mesures positives que je salue et que mon collègue Philippe Mouiller a eu l'occasion de mentionner tout à l'heure. Monsieur le ministre, au lieu de faire des chèques sans provision, comme le font les gouvernements depuis des années, le groupe Les Républicains veut muscler le texte avec des mesures pérennes, des mesures qui améliorent le pouvoir d'achat des Français, des salariés et des entreprises, et, surtout, des mesures d'économie,

les émissions carbone seront compensées. Nous demandons bien aux salariés de la centrale à charbon de Saint-Avold, sur la base du volontariat, de participer à cette relance dans des conditions que l'article 15

L'échéance a aussi été pensée pour être compatible avec le projet de compte épargne temps universel. Gardons donc aussi en tête la possibilité d'avancer sur certains chantiers.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

le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est parvenue à l'adoption d'un texte commun.